La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du vendredi 17 mai 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation

près de 100 000 élèves sortent chaque année du système éducatif sans formation ni diplôme ; le chômage des jeunes s'élève à 20 % ; notre pays occupe une place médiocre dans les classements internationaux et, malgré les réformes successives, cette place continue de se dégrader. Les dépenses pour l'éducation étant plus élevées que la moyenne des pays comparables, c'est non la question d'un manque de moyens qui se pose, mais Nous battons tous les records de reproduction des inégalités sociales et territoriales en matière éducative. Ainsi, 48 % des décrocheurs sont des enfants d'ouvriers, faute de bouclier de sécurité. Nous savons aussi que la grande majorité des élèves des filières professionnelles sont issus d'un milieu défavorisé. L'éducation nationale continue d'affecter et de rémunérer les enseignants en fonction plus de l'ancienneté que des besoins. Les directeurs d'école primaire ne disposent pas du statut et parfois des moyens nécessaires à leur mission. L'accroissement des charges administratives et les fréquents conflits entre enseignants et familles entravent les inspecteurs dans leur tâche et les empêchent de mener à bien leur mission pédagogique.

C'est d'autant plus préoccupant que, dans de nombreux territoires en difficulté, les enseignants font aujourd'hui partie des rares relais entre les citoyens et leurs institutions. À notre époque en proie au doute, à la défiance, au repli identitaire, où l'intelligence et la connaissance cèdent trop souvent le pas au délire et à l'ignorance, où la violence n'est jamais loin, à l'école, dans la rue ou sur les réseaux antisociaux- ce n'est pas un lapsus

! Au moins celui-ci a-t-il permis, au gré des discussions à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, que de nombreuses questions soient soulevées : inégalités sociales et territoriales, évaluation de l'école, maillage territorial, mixité, laïcité, santé, inclusion ou encore lutte contre le harcèlement. Si notre système éducatif concentre autant de problématiques différentes, c'est qu'il touche à ce que la République a de plus précieux : son avenir. C'est aussi la raison pour laquelle ce projet de loi a soulevé un certain nombre d'inquiétudes. Je voudrais saluer d'abord l'excellent travail de notre rapporteur, Max Brisson, qui a permis d'en dissiper plusieurs, ensuite votre attitude ouverte, monsieur le ministre, qui a permis un débat courtois et dépassionné, enfin l'implication de l'ensemble de nos collègues, qui ont siégé nuit et jour pour améliorer le texte et défendre leurs idées. Sans surprise, le Sénat a approuvé l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire, tout en offrant davantage de souplesse à son application. Nous espérons que cette mesure, associée à l'obligation de formation de 16 à 18 ans, sera un réel levier d'action contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes. Des mesures importantes ont été adoptées en matière d'engagement de la communauté éducative, du renforcement de l'école inclusive, de l'innovation pédagogique, de la formation des enseignants, de l'évaluation, de la gestion des ressources humaines. D'autres mesures importantes visent à renforcer la transmission et le respect des valeurs de la République en milieu scolaire. Pour prévenir les dérives, le Sénat a également adopté une disposition du Gouvernement visant à renforcer les sanctions contre les écoles privées hors contrat dont les activités ou le fonctionnement risqueraient de troubler l'ordre public. L'école est de plus en plus souvent victime des dérives communautaristes. Nous devons apporter une réponse claire et ferme à toute tentative d'endoctrinement. Il n'y a pas de place en France pour les écoles pratiquant l'éducation à la haine dans le plus grand mépris des valeurs de la République. Après un débat de haute tenue, bien éloigné des polémiques qui l'ont précédé, la Haute Assemblée a supprimé la possibilité de fusionner écoles et collèges au sein d'un établissement public local. Cette mesure suscitait de l'inquiétude parmi les élus locaux, en particulier les maires ruraux, et la communauté éducative concernée. Nous avons fait le constat qu'une telle réforme de l'organisation de l'école ne pouvait se faire par voie d'amendement, sans étude d'impact et sans concertation préalable avec l'ensemble des acteurs concernés. Nous ne pouvons qu'espérer que les débats qui se sont tenus sur ce sujet, notamment sur l'initiative de notre collègue Jacques Grosperrin, ne resteront pas lettre morte. pour conclure, Hannah Arendt : « C'est [ ...] avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer à la tâche de renouveler un monde commun. » Le projet de loi que nous avons examiné n'est pas la panacée à tous les maux qui touchent, dès l'aurore, notre société. par exemple abordé ni la question de la modernisation des méthodes pédagogiques, ni la valorisation du métier d'enseignant, ni la crise d'autorité qui touche autant l'école que l'État. Il me semble pourtant que ce texte va dans le bon sens et que la contribution du Sénat l'a substantiellement enrichi. Notre groupe votera donc ce projet de loi. La parole

L'affirmation de divers principes, des mesures juxtaposées ou ajoutées en cours de lecture forment un ensemble qui ne traitera malheureusement pas les travers de notre système éducatif, dénoncé régulièrement par les études comme inégalitaire et peu performant. Lors des débats, monsieur le ministre, vous avez dit qu'aux deux extrémités de notre système le projet de loi apportait « deux acquis fondamentaux » : l'obligation d'instruction abaissée à 3 ans et la formation obligatoire de 16 à 18 ans. Cependant, ces deux mesures ont surtout valeur de symbole, tout comme l'intitulé de ce projet de loi « pour une école de la confiance ». Je ne ferai pas preuve d'originalité en rappelant que la quasi-totalité des enfants sont déjà scolarisés à l'âge de 3 ans. À l'autre extrémité du système, assurer que les jeunes de 16 à 18 ans devront être en formation et tenter d'identifier ceux qui ne le sont pas ne règle malheureusement pas le problème de la déscolarisation.

au lieu de rassembler, ce projet de loi a failli désunir. Ces derniers mois, loin de la confiance souhaitée, il a soulevé l'inquiétude, voire l'opposition de la communauté éducative, des parents et des élus locaux. Le Sénat s'est donc employé à retrouver l'apaisement.

Le Sénat est intervenu tout d'abord pour combler les lacunes du texte. Je pense notamment à la mise en oeuvre de la scolarisation à 3 ans : les besoins de compensation des communes n'avaient pas été entièrement pris en compte, la situation des jardins d'enfants non plus. La fatigue de l'enfant devait être prise en considération au moyen d'assouplissements. La mesure phare du projet de loi nécessitait finalement divers ajustements. Je pense également au chapitre entier introduit par l'Assemblée nationale sur l'école inclusive, qui appelait de nombreuses précisions. Le Sénat est également venu apporter des garde-fous à certaines dispositions controversées.

Sur le plan des symboles, le Sénat a tenu à réaffirmer l'autorité des enseignants et des directeurs et le respect qui leur est dû, à un moment où les agressions, verbales et physiques, n'ont jamais été aussi nombreuses. Le choix des symboles, dans un texte sur l'école, est important et nous tenions à ce que chacun se sente soutenu. Nous avons également maintenu la présence de symboles républicains dans les classes, comme l'avaient souhaité les députés, et nous avons réaffirmé l'importance du principe de laïcité. Notre rapporteur a introduit des sujets importants qui ne figuraient pas dans le projet de loi, mais sur lesquels nous appelions à légiférer de longue date : le statut du directeur d'école ou la formation continue des enseignants, qui sont des éléments clés pour améliorer la qualité de l'enseignement en France. Enfin, le Sénat a entendu la demande des élus locaux, de la communauté éducative et des parents en supprimant l'article 6, qui a fait grand bruit en étant introduit sans concertation préalable à l'Assemblée nationale. Les fameux établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux, regroupant écoles et collèges, sont apparus en cours de procédure sans qu'il y ait eu ni débat préalable, ni étude d'impact, ni avis du Conseil d'État. Or la concertation et l'analyse sont des préalables indispensables pour introduire des mesures nouvelles. La polémique qui a eu lieu et qui n'est pas de votre fait, monsieur le ministre, est regrettable. Sur certains territoires, l'idée répond à un réel besoin, comme le montrent les témoignages d'élus expérimentant actuellement ces regroupements. ces regroupements. Le dispositif proposé était perfectible, ce que j'ai pu démontrer, ainsi que plusieurs de mes collègues, en proposant une réécriture donnant toute l'initiative aux élus, associant la communauté éducative et en les assurant par la loi du maintien des écoles dans chaque village ainsi que des fonctions de directeur. semblé que la priorité était de sortir du cercle de défiance que l'article avait suscité. Une telle mesure ne pouvait se décréter sans dialogue de fond, alors que de fortes inquiétudes s'étaient exprimées. Vous avez vous-même conclu en séance, monsieur le ministre- je vous en remercie -, à la nécessité d'ouvrir maintenant une concertation sur le sujet. Nous espérons que tel sera le cas et que les députés se joindront à nous sur ce point. Nous appelons également de nos voeux un accord en commission mixte paritaire concernant les nombreux ajouts, précisions et modifications que nous avons introduits. La rédaction issue du Sénat est équilibrée, aboutie et repose sur le dialogue. Je conclurai mon propos par un extrait du discours d'investiture au Sénat du président Jules Ferry, le 27 février 1893-

N'est-ce pas précisément l'état d'esprit de cette grande Assemblée, ce qui donne à vos débats tant de noblesse, ce qui assure ici aux relations personnelles tant de charme et de dignité ?

qui aura permis à chaque groupe de défendre ses propositions sur l'école, de confronter ses points de vue, d'argumenter- parfois avec passion, mais toujours dans un climat digne et serein qui fait honneur à la Haute Assemblée. La bonne tenue de ce débat a été rendue possible par votre souci permanent, monsieur le ministre, d'expliquer et de clarifier chacun de vos choix. En effet, c'est toujours dans l'écoute et le dialogue que vous avez discuté avec les sénateurs et ceux-ci ont, je pense, apprécié la qualité et la franchise de vos réponses.

Nous l'avons dit, ce projet de loi n'a pas vocation à répondre seul aux défis de l'école : d'abord parce que tout ne relève pas de la loi en cette matière si spécifique qu'est l'éducation nationale, parce que ce texte s'inscrit dans une politique plus ambitieuse en faveur de l'élévation du niveau général des élèves et d'une plus grande justice sociale. Ce projet de loi, parfois jugé hétéroclite et secondaire, aura permis des débats nourris sur des enjeux fondamentaux, loin d'être symboliques. École inclusive, décrochage scolaire, mixité sociale, langues régionales, statut des directeurs d'école ou encore formation des enseignants : personne ne me contredira si je dis ici que nos échanges ont été denses et souvent teintés de la passion des anciens maires et des enseignants qui composent cette maison. Au cours de la discussion, le projet de loi a donné lieu à de nombreux points d'accord ainsi qu'à certaines clarifications attendues. J'espère, monsieur le ministre, que le Gouvernement en tiendra compte pour la suite du débat, dans le respect du bicamérisme. Je pense d'abord à l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire, votée à l'unanimité par notre Assemblée. Loin d'être accessoire, cette mesure consolide le cadre de l'école républicaine. J'ai rappelé l'immense défi que cela provoquerait dans certains territoires, notamment à Mayotte et en Guyane. Le Sénat y a été très sensible et a adopté une expérimentation consistant à faciliter les constructions scolaires. je pense aussi aux mesures profondément sociales que constituent l'obligation de formation de 16 à 18 ans, le renforcement de l'école inclusive ou encore le prérecrutement. Je pense également à l'article 1, qui, loin d'être un instrument pour museler les enseignants, rappelle ce qui fonde la relation entre le maître et l'élève. aux établissements publics d'enseignement des savoirs fondamentaux pour lesquels, avec votre assentiment, monsieur le ministre, le Sénat a adopté, sans s'opposer radicalement au principe, une position de sagesse afin de privilégier un dialogue concerté avec l'ensemble de parties prenantes. Des divergences demeurent nécessairement dans pareil exercice et nous regrettons de ne pas avoir convaincu notre assemblée sur d'autres points. C'est le cas de l'accompagnement financier prévu en faveur des communes lié à l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire Le Sénat a adopté un mécanisme de régulation au profit des communes ayant déjà fait le choix de participer à la prise en charge des dépenses relatives aux classes maternelles privées. S'il nous semble indispensable que l'État s'engage sur les nouvelles dépenses, il ne saurait compenser dans une forme de rétroactivité celles qui étaient déjà engagées par le passé au titre de la libre administration des collectivités territoriales. constat est identique concernant la dérogation accordée aux jardins d'enfants. Il est assez surprenant d'observer qu'avant l'examen au Sénat le Gouvernement a été injustement accusé de sonner le glas de l'école maternelle au profit des jardins d'enfants pour se voir finalement reprocher l'exact opposé dans cet hémicycle. Ce n'est pas vrai ! À l'arrivée, le Sénat a choisi de pérenniser la dérogation accordée à ces structures. Nous respectons ce choix, comme nous respectons le travail qui a été réalisé. Toutefois, l'esprit de cette loi étant de renforcer l'école maternelle comme socle de l'école républicaine, nous restons convaincus qu'il eût été préférable de limiter cette dérogation dans le temps pour accompagner les jardins d'enfants vers une évolution. Nous regrettons enfin de ne pas avoir convaincu le Sénat sur le statut des directeurs d'école. En souhaitant envoyer un signal, certes positif dans l'élaboration d'un véritable statut, la majorité sénatoriale risque d'entraver le dialogue social en créant de la défiance parmi le corps enseignant. En effet, la question du lien hiérarchique, notamment de l'évaluation, est loin de faire l'unanimité parmi les directeurs eux-mêmes. À cet égard, notre groupe réitère son souhait de voir le statut du directeur d'école faire l'objet d'une concertation avec les syndicats. Cela étant, notre vote sera déterminé par des choix nettement plus regrettables, auxquels nous ne saurions souscrire. Je pense d'abord à l'interdiction du voile pour les sorties scolaires,

Appliquée de 2010 à 2013, cette mesure a déjà démontré son caractère particulièrement injuste et inefficace. Là encore, dans un texte appelant à la confiance entre la communauté éducative, les parents et les élèves, ces mesures jettent l'anathème sur une partie des familles, au risque de creuser plus encore les inégalités. En définitive, le Sénat a largement adopté les principales dispositions de ce projet de loi, parce que celles-ci vont dans le bon sens. Cependant, malgré d'évidentes clarifications, nous devons nous prononcer sur un texte qui comporte également des mesures qui contreviennent, selon nous, à son ambition sociale.

à Mme Céline Brulin, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà plusieurs semaines que nous débattons, ici, au Sénat, du devenir de notre système éducatif, alors que dans le pays résonnent inquiétudes et colère. C'est une très bonne chose que les parents d'élèves, les élus locaux, évidemment les enseignants, et, finalement, toute la société se soient ainsi mêlés du débat. L'école concentre toutes les exigences d'égalité, de justice sociale et même d'ascenseur social, qui continuent de mobiliser le peuple français malgré les offensives libérales nous sommant d'abandonner cette promesse républicaine. Cette mobilisation n'est pas étrangère à l'abandon des « établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux » regroupant écoles et collèges. Nous nous en félicitons, mais nous resterons vigilants face à toutes les tentatives de prendre appui sur d'éventuels intérêts pédagogiques pour accélérer la désertification scolaire dans nos territoires, car la proximité et l'égalité d'accès sont pour nous des principes fondateurs de notre système éducatif. Là s'arrêtent malheureusement nos motifs de satisfaction. Beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, aviez pris l'engagement que nos débats soient à la hauteur de l'enjeu, l'école de la République méritant mieux que des postures. Cet objectif a parfois été manqué, et de beaucoup : considérer, par exemple, que la suspension des allocations familiales réglera l'absentéisme, c'est être bien loin de la responsabilité qui est la nôtre Cette mesure, et chacun le sait ici car elle a été expérimentée, est aussi injuste que contre-productive. Très bien ! Ce n'est pas vrai ! Il est regrettable, et pour tout dire assez honteux, que de tels errements idéologiques aient eu leur place dans notre assemblée. Qui peut vraiment croire qu'appauvrir les familles, tout particulièrement celles qui rencontrent des difficultés sociales et éducatives, serait la solution aux problèmes de l'école ? Ce n'est malheureusement pas la seule mesure, introduite par votre majorité sénatoriale, que nous ayons à regretter. Je pense à l'annualisation du temps de service des enseignants ou à leur formation continue « en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement ». Dans le droit-fil de votre choix, de porter de un à trois le nombre de jours de carence dans la fonction publique en cas de maladie. J'ai encore en mémoire ces enseignants victimes de violences, auditionnés en commission, qui avaient clairement mis en accusation cette décision, la jugeant précisément violente. « Vous avez décidé de nous retirer 250 euros de salaire parce que, enseignant à plusieurs dizaines d'élèves chaque semaine, il y a peu de chances que nous échappions à l'épidémie de gastro-entérite cet hiver », nous avaient-ils dit en substance. Là encore, qui peut croire que nous répondrons ainsi à la crise de recrutement que nous connaissons dans l'enseignement ? Au-delà, c'est le coeur du texte qui demeure le principal problème : notre système scolaire à deux vitesses ne répond aucunement au véritable enjeu, qui est d'en finir avec la reproduction des inégalités ; au contraire, il risque de les aggraver. Après avoir réalisé la massification de l'enseignement, c'est à sa démocratisation que la France devrait s'attaquer. Voilà qui serait de nature à restaurer la confiance. Les établissements publics locaux d'enseignement international, qui n'ont d'ailleurs de public que le nom puisqu'ils pourront être financés par des dons privés, continuent par exemple, malgré les correctifs cosmétiques qui leur ont été apportés, d'entériner une logique profondément inégalitaire. Le remplacement du Cnesco par un conseil d'évaluation de l'école, qui généralisera la mise en concurrence des établissements, par l'évaluation, vise les mêmes objectifs. Nos craintes concernant le recours aux assistants d'éducation, notamment pour les remplacements de courtes durées, dans les zones les plus déficitaires, souvent les quartiers populaires ou les zones rurales, ne sont pas non plus dissipées.

Le sort réservé à l'école inclusive tourne encore plus explicitement le dos aux valeurs de l'école publique. La mise en place des pôles inclusifs d'accompagnement localisés,

Nous n'avons malheureusement pas pu approfondir la question de la situation des accompagnants de ces enfants, la plupart de nos amendements ayant malheureusement été déclarés irrecevables.

maintenant l'article 1 du texte, qui demeure toujours aussi dangereux pour l'exercice de la citoyenneté des professeurs. Fonctionnaires, bien évidemment soumis à des devoirs, ceux-ci n'en sont pas moins des citoyens, qui ont d'ailleurs pour mission de former d'autres citoyens, de futurs citoyens. Les procédures disciplinaires qui se multiplient actuellement ne sont évidemment pas faites pour nous rassurer sur ce point non plus. Nous resterons vigilants pour empêcher que des dispositions rejetées ou supprimées soient réintroduites par voie réglementaire, comme il est bien trop souvent possible de le faire en matière d'éducation. Notre groupe votera contre ce texte, qui suscite toujours, avec raison, la défiance parmi les parents d'élèves, les enseignants, les élus locaux et tous ceux qui sont attachés à l'idéal de l'école républicaine. Nous avons la conviction

La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour le groupe socialiste et républicain.

bonne chance ! Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quel marathon législatif avons-nous vécu la semaine dernière ! Les débats ont été riches, intenses, parfois passionnés, mais l'objet et les enjeux de ce texte de loi le valaient bien. Ils ont démontré, une fois de plus, l'importance du bicamérisme : l'apport du Sénat est crucial pour alimenter le travail parlementaire, l'enrichir et permettre une forme de maturation nécessaire à l'ouvrage législatif, dans le respect de toutes les sensibilités. Je tiens à saluer mes collègues chefs de file Maryvonne Blondin, Claudine Lepage et Maurice Antiste, qui ont porté notre parole avec compétence et conviction pour l'école républicaine. Monsieur le ministre, nous n'avons pas la même vision de l'école de la République. Au fil de l'examen de ce texte, si vous avez semblé être à l'écoute, vous ne nous avez pas entendus sur plusieurs points, et nous le regrettons. Sur de nombreuses mesures, le temps d'étude préalable a été trop réduit. La concertation a manqué. Le projet de loi est examiné en procédure accélérée afin de pouvoir être appliqué à la rentrée par voie de décrets et d'ordonnances. Cet empressement n'est pas compatible avec le temps long nécessaire à toute réforme de l'éducation. Je veux toutefois souligner un réel point positif : l'abandon des établissements publics locaux Ces EPLESF risquaient d'entraîner des bouleversements profonds dans la structure du système scolaire et auraient eu lourdes conséquences pour les élèves, leurs familles, les personnels et les territoires, notamment ruraux. Cette suppression est une victoire pour tous les acteurs de la communauté éducative et les élus, qui s'étaient fortement mobilisés contre ces

Nous sommes aussi satisfaits que le Gouvernement, conformément à l'engagement pris le 8 février à Rennes, ait apporté son soutien à l'article 6 A, qui traduit les conclusions de la conférence territoriale de l'action Sur l'article 4, nous nous réjouissons que la commission ait ouvert la compensation à toutes les communes, même s'il est dommage que les amendements que nous avons portés, lesquels visaient à apporter davantage de garanties sur leurs dépenses nouvelles, aient été rejetés. Au-delà de ces quelques points, l'esprit général du texte n'a pas changé. Nos inquiétudes concernant l'article 8, sur l'annualisation des heures et l'orientation des élèves, n'ont pas été entendues. Les expérimentations peuvent parfois permettre de belles avancées, mais elles ne doivent pas se faire au détriment des élèves. L'article 6 confie une autorité hiérarchique aux directeurs d'école. Nous l'avons dit, ce n'est pas en divisant l'équipe éducative que l'on renforcera sa cohésion ou l'autorité de ses membres.

qu'il ne s'agit pas là de compenser la pénurie d'enseignants dans certains territoires ou certaines matières ni de créer une sous-catégorie de professionnels. Ce projet de loi aurait dû améliorer les conditions de travail des personnels, mais ce n'est, hélas ! pas le cas. La majorité sénatoriale a aggravé encore leur situation en allant plus loin que le Gouvernement. Elle a ainsi prévu l'obligation de formation continue « en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement » et rejeté les garde-fous que nous avions proposés. Je ne peux passer à côté de l'article 1, dont la rédaction continue de faire planer la suspicion sur l'ensemble des membres de la communauté éducative.

Nous ne comprenons pas non plus l'obstination à vouloir supprimer le Cnesco, car cette instance fonctionne bien. En mettant en avant les travaux de la recherche scientifique sur les politiques éducatives, elle permet de sortir de débats souvent stériles. Les quelques modifications apportées, pour augmenter la part des parlementaires dans la composition de votre nouveau conseil, monsieur le ministre, ne changent pas grand-chose sur le fond. Finalement, l'examen de ce texte au Sénat a surtout mis en évidence, si certains doutaient encore de son existence, le clivage gauche-droite. Le texte qui ressort de nos travaux s'éloigne davantage de nos valeurs d'égalité et de justice sociale et de ce que nous pouvions attendre d'un texte sur l'école républicaine face aux enjeux du XXI siècle. Les vieux serpents de mer de la droite ont ponctué les débats, comme l'interdiction des signes religieux ostentatoires pour les accompagnateurs ou accompagnatrices lors des sorties scolaires, ou encore la suppression des allocations familiales pour les parents d'élèves absentéistes. Cette mesure, que nous avions supprimée en 2013,

Pourtant, ce texte aurait pu sortir du Sénat avec une vision plus progressiste et plus sociale. Nous avons tout fait pour, en déposant de nombreux amendements. Certains, retoqués au titre des articles 40 et 45 de la Constitution, portaient sur l'université. À ce sujet, je souhaite évoquer les récents dysfonctionnements de Parcoursup, qui nous alertent sur les failles de cette plateforme et qui plongent des milliers de lycéens dans l'angoisse et l'incertitude. Pour en revenir à nos amendements,

Vous avez ainsi choisi de rejeter la suppression des PIAL, qui constituent un simple outil de gestion comptable et de mutualisation des AESH, et non un dispositif permettant de cibler les besoins des enfants et d'accroître la qualité de leur accompagnement. également choisi de rejeter la sensibilisation des élèves aux violences faites aux femmes et la lutte contre les violences sexistes, dans le primaire et le secondaire. Vous avez de même choisi de rejeter nos amendements visant à décharger les missions locales de nouvelles obligations, alors que leur situation financière reste délicate.

En conclusion, ce sont deux droites qui se rejoignent autour d'une même vision de l'éducation, plus libérale. Pour le groupe socialiste, ce texte comprend bien trop de mesures déstructurant le cadre national de l'éducation. le cadre national de l'éducation. Nous voterons contre ce texte, car nous sommes de celles et ceux qui croient en une école émancipatrice, en une école où l'on devient d'abord un citoyen ou une citoyenne accompli, soucieux de l'intérêt collectif pour se préparer à un emploi, en une école qui permette de se construire, peu importe d'où l'on vient : une école de la République ! La parole est à Mme Françoise Laborde, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Le manque de concertation, dénoncé par la communauté éducative, a été doublé d'une forme de précipitation, le tout aboutissant à un texte aux dispositions trop diverses. loi aurait gagné en force, et je l'ai déjà dit, à rester centré sur son objectif de départ : rendre obligatoire la scolarisation des enfants dès l'âge Je vous l'accorde, notre système éducatif a besoin de confiance, celle des Français envers les enseignants, celle du monde éducatif en sa propre capacité à relever les défis, et enfin celle des collectivités territoriales. Or les sénateurs du groupe du RDSE sont inquiets concernant l'égal accès des élèves à l'instruction sur l'ensemble du territoire. Ce doute n'a malheureusement pas été levé

Le vote d'un amendement à l'article 1, visant à inscrire dans la loi le rôle de l'école dans la transmission des valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, était était nécessaire, bien qu'insuffisant face aux défis auxquels elle est confrontée sur le terrain social, territorial, mais aussi technologique. Construire l'école de la confiance, c'est d'abord s'appuyer sur des enseignants

Les apports du Sénat à ce texte s'agissant des ressources humaines de l'éducation nationale sont indéniables. Je salue l'adoption de la formation continuée et de la formation continue pour tous les professeurs du premier comme du second degré, mesures permettant de rendre le métier d'enseignant plus adapté et qu'il faudra pouvoir conserver en commission mixte paritaire. La sensibilisation des futurs professeurs aux enjeux de l'environnement et du respect de la biodiversité, apport auquel le groupe du RDSE a contribué, était urgente afin qu'ils intègrent à leur tour ces sujets, encore trop rarement dispensés, Si j'approuve l'évolution de la maquette de formation des Inspé- eh oui ! -vers l'usage des outils et ressources numériques en classe, je regrette que mon amendement visant à donner la priorité à l'utilisation de logiciels libres dans le service public de l'enseignement n'ait pas pu être discuté, alors que le lien m'apparaît pourtant limpide avec le texte en discussion. Nous avons entendu, monsieur le ministre, vos engagements sur la réforme du prérecrutement des futurs enseignants, qui va dans le bon sens en assurant leur formation sur le terrain. Nous serons attentifs à ce que ce dispositif ne soit pas dévoyé. Le statut d'assistant d'éducation, ouvert aux étudiants de L2, ne saurait être un moyen de remplacer des titulaires. Permettez-moi d'évoquer d'autres points de la discussion qui nous ont semblé significatifs et sur lesquels nous serons vigilants. Nous sommes opposés aux établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux proposés à l'article 6 . La suppression de cet article avait été adoptée unanimement en commission, l'amendement de notre collègue Grosperrin nous ayant permis d'engager une discussion de fond dans l'hémicycle, avant son retrait. J'espère, monsieur le ministre, que vous veillerez à ce que cet article ne revienne pas. Concernant l'école inclusive, je me félicite de ce que le Sénat ait inscrit la formation continue des AESH dans le texte, reconnaissant ainsi leur rôle à part entière dans l'équipe éducative et le besoin de renforcement de leur professionnalisation. Toutefois, j'estime que le texte n'est pas encore satisfaisant sur les PIAL. Ces pôles peuvent être utiles, à la condition que leur création résulte d'une concertation organisée entre l'éducation nationale, le champ médico-social et les collectivités territoriales, afin de s'insérer dans un espace géographique pertinent et en nombre adapté dans le département. Il faut laisser plus de place à la concertation entre les acteurs. Notre groupe approuve l'obligation de formation professionnelle de 16 à 18 ans, à condition de s'appuyer sur le réseau du service public de l'orientation tout au long de la vie. Tel est le sens de l'un de nos amendements qui Concernant le statut des directeurs d'école, le résultat est en deçà de nos espérances, car une simple participation aux évaluations ne suffira pas à rendre la fonction plus attractive ou plus légitime au sein de l'établissement. Quant aux établissements privés hors contrat, des dispositions bienvenues ont été adoptées pour compléter la loi Gatel. Il s'agit de l'obligation de déclarer le changement de projet d'établissement ou d'objet d'enseignement et la création d'une nouvelle sanction, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de non-respect des mises en demeure. Je regrette la création du conseil d'évaluation de l'école, en lieu et place du Cnesco, qui permettait une évaluation indépendante, avec un volet recherche scientifique très important. L'un aurait pu être complémentaire de l'autre. Il est fort dommage ce projet de loi n'ait pas été l'occasion d'aborder la question de la visite médicale du personnel enseignant. Nous nous mobiliserons de nouveau sur cette problématique lors de l'examen En ce qui concerne la santé des élèves, le dispositif prévu est encore un peu décevant. Mais nous avons pu faire voter le maintien de l'autonomie des infirmiers scolaires. Nous approuvons par ailleurs l'autorisation donnée au médecin scolaire de prescrire certains actes et produits de santé. Nous sommes fortement opposés au contrat de responsabilisation transposant les dispositions Ciotti sur la suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme de l'élève, car nous considérons que c'est une double peine qui fragilise les plus vulnérables et renforce le rejet de l'école. Nous avons débattu de l'interdiction du port de signes, ou tenues, par lesquels se manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, étendue aux sorties scolaires et aux personnes concourant au service public de l'éducation. Une majorité de notre groupe a voté en faveur de cette mesure, qui ne survivra peut-être pas en En conclusion, je tiens à souligner les apports majeurs du Sénat sur le métier d'enseignant, qui manquaient cruellement à ce texte pour renouer avec la confiance en l'école. Malgré tout, nombre de mes collègues du groupe du RDSE jugent le texte déséquilibré, les enjeux liés à l'école dans les territoires étant pris en compte de manière bien trop parcellaire. L'école est parfois le dernier service public. Nos élus attendent une politique de l'école dans les territoires qui, au vu de ce texte, reste encore à inventer. Telles sont les raisons pour lesquelles une large part de notre groupe s'abstiendra.

préparatoire et près d'une semaine de discussions, parfois passionnées, dans cet hémicycle. Le vote de ce texte marque l'aboutissement d'un important travail, en commission comme sur le terrain, dans un climat qui n'a pas toujours été des plus sereins, en tout cas à l'extérieur de la Haute Assemblée. À l'issue de ces quatre jours de séance, nous sommes convaincus que ce texte a évolué grâce aux apports du Sénat. Il était grand temps de dépassionner le débat en prenant en compte, dans nos propositions, le point de vue des acteurs locaux, des élus, des personnels de l'éducation et des parents. C'est en procédant de la sorte que le changement est possible en matière éducative, mais cela nécessite du temps, de l'expérimentation et l'association étroite des différents acteurs. je tiens à saluer l'écoute dont vous avez fait preuve pendant nos débats et la qualité de nos échanges tout au long de nos travaux. Si nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout, nous espérons néanmoins que vous saurez reconnaître les apports du Sénat à ce texte important. Je souhaite également remercier de nouveau le rapporteur, Max Brisson, et la présidente de la commission, Catherine Morin-Desailly, pour leur implication dans la conduite de nos débats. C'est le vif attachement que nous portons, toutes et tous, à l'école de la République qui a conduit nos réflexions et, nous l'espérons, permis d'améliorer ce projet de loi de manière constructive constructive et approfondie. Sans bien entendu mettre de côté nos problématiques locales ni les sujets qui nous tiennent personnellement à coeur, nous pouvons dire que nous avons ici travaillé en ayant ayant à l'esprit l'intérêt des générations futures. Faire que chaque enfant, quelle que soit sa situation, puisse trouver sa place à l'école : voilà ce qui a guidé nos travaux. Il a pu être reproché au projet de loi tel que nous l'avons reçu de l'Assemblée nationale de manquer d'un certain souffle, de ne pas contenir de dispositions véritablement à même d'apporter des réponses aux enjeux auxquels fait face notre système scolaire, ou encore d'être finalement un texte un peu fourre-tout. C'est heureux que le groupe que je représente ait pu vous convaincre d'enrichir le texte qui nous était soumis sur plusieurs points importants. À titre d'exemples, pour n'en donner que quelques-uns, l'éducation au développement durable et à la protection de l'environnement a notamment été consacrée dans notre droit, l'initiative de notre collègue le président Hervé Maurey. De même, l'autonomie des infirmiers scolaires a été défendue grâce à notre collègue Jocelyne Guidez. Grâce à la présidente Catherine Morin-Desailly, la formation des professeurs sera structurée par la maîtrise des outils et des ressources numériques. Je tiens également à citer nos avancées d'une meilleure implication des territoires et des élus locaux, avec une prise en compte réelle de la dimension territoriale des inégalités dans la répartition des moyens du service public de l'éducation ou encore avec une meilleure association des communes dans l'élaboration des conventions de formation continue des professionnels intervenant auprès des enfants de moins de 6 ans. D'autres dispositions, que nous avons soutenues, doivent également être mises en lumière. Je pense aux compromis trouvés sur l'annualisation du temps de travail, sur les jardins d'enfants ou sur les visites médicales, à la lutte contre le prosélytisme, à la lutte contre l'absentéisme par la possibilité de retenues sur les allocations familiales versées aux parents d'élèves de moins de 16 ans, à l'ensemble des mesures en faveur de l'école inclusive, aux contractualisations rendues possibles avec les établissements privés sous contrat afin d'encourager la mixité sociale, ou encore aux solutions pour répondre aux problèmes de recrutement, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, avec l'ouverture des postes à profil. Vous aurez constaté, monsieur le ministre, notre profond attachement à ce que, à l'avenir, davantage d'initiatives soient laissées aux acteurs locaux, aux élus, aux personnels de l'éducation, aux parents, pour trouver les solutions et les moyens de répondre aux besoins des territoires en matière d'éducation. Mon groupe et moi-même souhaitons vivement que ces améliorations sensibles sauront convaincre nos collègues de l'Assemblée nationale lors de la commission mixte paritaire. Je reviendrai un instant sur la disposition qui a été, de loin,

Si les discussions ont été aussi animées que les semaines de mobilisation le laissaient prévoir, nous avons, il me semble, réussi à sortir par le haut de cette situation. Nous comptons désormais sur votre sagesse, monsieur le ministre, pour que l'école du socle fasse l'objet d'un véritable travail approfondi, dans un climat apaisé et à même de satisfaire les différentes parties prenantes de notre système scolaire, toujours dans l'intérêt des élèves. Le groupe Union Centriste prendra toute sa part à ce travail, comme aux réflexions plus larges sur l'avenir de notre école. La restitution prochaine des travaux de la mission d'information sur les nouveaux territoires de l'éducation sera ainsi l'occasion d'enrichir le débat de nouvelles propositions, comme les résultats de la mission Mathiot-Azéma, que nous analyserons avec attention, bien entendu. Pour conclure, épargnons-nous ici les descriptions apocalyptiques sur la situation de notre système scolaire, les « condoléances aux futurs illettrés », les rapports savants sur l'échec scolaire, ou encore la dénonciation des « usines à cancres ». Non pas que la critique soit toujours inutile, mais ce qui aura compté tout au long de nos travaux, c'est moins le diagnostic que les remèdes. Le groupe Union Centriste votera ce texte ainsi amendé par notre assemblée. Mes collègues et moi-même resterons bien sûr attentifs à sa mise en oeuvre ; nous veillerons à toujours défendre notre école républicaine, celle qui sait intégrer, celle qui fait du mérite- et non de l'argent ou des relations -le véritable facteur de la promotion sociale. Jules Ferry s'était fait un serment : l'éducation du peuple. Cette ambition a inspiré l'école du brassage social et de la promotion individuelle. Cet idéal reste d'actualité, même si les moyens de l'atteindre ont changé. L'école doit avoir plus que jamais l'ambition de donner à chacun sa chance.

nos collègues Daniel Dubois, Dominique de Legge et Patricia Schillinger, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Je rappelle qu'une seule délégation de vote est

Merci,

Plusieurs milliers de candidats qui avaient reçu une réponse favorable de Parcoursup le soir se sont réveillés avec un avis négatif le matin ... Madame la ministre, vous expliquez ce dysfonctionnement, qui toucherait 7 % des candidats, par un problème informatique.

pourquoi faire porter aux établissements la responsabilité d'un revirement qui est la conséquence de décisions politiques que vous n'assumez pas ? Exactement ! En janvier, le Défenseur des droits vous avait demandé de rendre publics les critères de sélection des établissements et de réformer Parcoursup pour mettre fin aux discriminations subies par les lycéens des filières technologiques et professionnelles. Nous attendons toujours vos réponses à ces questions essentielles, madame la ministre

Le service qui permet de surveiller le fonctionnement de la plateforme a immédiatement relevé ces anomalies et les établissements eux-mêmes ont appelé le ministère pour signaler les erreurs et obtenir une aide pour les corriger.

Madame la ministre, je doute sincèrement que les candidats et les parents soient rassurés par la clarté de vos explications. Très bien En ce qui nous concerne, nous continuerons à dénoncer la violence de ce dispositif, qui, l'an passé, a éloigné de l'enseignement supérieur plus de 180 000 lycéens. Nous continuerons de défendre un enseignement supérieur accessible à tous les bacheliers, sans discrimination.

le 11 avril dernier, la justice reconnaissait Monsanto responsable du dommage causé à l'agriculteur Paul François, victime du Lasso, un puissant herbicide. Voilà quelques jours, aux États-Unis, Monsanto était de nouveau condamné à indemniser les victimes du Roundup. Depuis près de deux ans, le groupe socialiste du Sénat demande avec insistance la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytosanitaires et, depuis près de deux ans, le Gouvernement refuse cette création.

le scandale Monsanto et la découverte de pratiques de lobbying insupportables. Monsieur le ministre, pour toutes ces raisons, il est temps de sortir du déni politique et industriel, en faisant en sorte que les grandes firmes prennent et assument toutes leurs responsabilités. C'est comme cela aussi que nous changerons durablement les pratiques. Parce que les

vous le savez, ont déjà permis de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Avec François de Rugy, Frédérique Vidal et Didier Guillaume, j'ai installé officiellement le 10 avril dernier le comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national de réduction des produits phytosanitaires. S'agissant de la création du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, il convient d'être justes et attentifs à la souffrance des victimes. Il convient aussi d'être responsables en mettant en place un dispositif d'indemnisation cohérent avec les connaissances scientifiques

Lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale en janvier dernier, j'ai proposé que la discussion reprenne lors des débats sur les lois de finances ou lors de la poursuite de l'examen de la proposition de loi. J'ai pris l'engagement qu'y figurent des articles tendant à créer ce fonds, sur la base des discussions ayant eu lieu lors de l'examen de votre proposition de loi. En attendant, un rapport sur le financement et les modalités de création d'un fonds d'indemnisation doit vous être rendu

Quelques phrases de ce chef-d'oeuvre : « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs. Attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartelez-les pour passer le temps ... » Sur plainte du ministre de l'intérieur, ce grand artiste a été condamné ... à une amende avec sursis Dans ces conditions, pourquoi se priver ? Nick Conrad, c'est son nom, a donc récidivé ces jours-ci avec un nouvel opus d'aussi haut niveau : « Je baise la France jusqu'à l'agonie. Je brûle la France. J'vais poser une bombe sous son Panthéon. » À la fin du clip, il étrangle en gros plan une femme blanche. Le ministre de l'intérieur a porté plainte immédiatement. Il a eu raison. Mais avec la loi actuelle, l'auteur sera condamné dans deux ans à une peine légère. Entre-temps, le clip aura été vu quelques millions de fois. Le racisme n'est qu'une des plaies béantes des réseaux dits « sociaux », et le racisme anti-blanc n'est pas plus tolérable qu'un autre. Les autres plaies s'appellent sexisme, intimidation, usurpation d'identité, harcèlement, injures et menaces de mort. Les Gafa font le service minimum pour conserver leur business juteux. Mais Mark Zuckerberg a dû convenir lui-même qu'il n'avait pas les moyens de réguler efficacement ses plateformes et n'a rien trouvé de mieux que d'appeler les gouvernements à légiférer. Il est urgent de le prendre au mot. Les Allemands n'ont pas hésité à faire une loi ordonnant le retrait de contenus haineux sous vingt-quatre heures. Qu'attendons-nous pour les imiter ? Une proposition de loi est en préparation à l'Assemblée nationale, Je voudrais être sûr, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement ne l'accueillera pas d'une main tremblante. Il ne s'agit pas de liberté d'opinion ni de censure, mais de lutte contre des délits graves, le plus souvent commis anonymement. Il me semble même que le sujet est tellement grave qu'il justifierait un débat national et une unité européenne aujourd'hui balbutiante. La haine ou le racisme n'ont pas leur place chez nous. Nous ne sommes pas au Far West et, même dans la jungle, il y a une loi. Il est urgent de faire respecter les nôtres

je voudrais évoquer avec vous la situation de Vincent Lambert et le débat, comme l'émoi, qu'elle suscite dans le pays. Je voudrais le faire sans céder à la tentation qui, dans cette affaire, peut tous nous guetter, quelles que soient nos convictions intimes, celle des postures établies d'avance, des certitudes toutes faites. Devant une telle situation, ayons l'humanité de compatir et l'humilité de reconnaître. Compatir, parce qu'au-delà des positions des uns ou des autres il y a un drame ; il y a le silence d'un homme ; il y a la douleur déchirante d'une famille déchirée, exposée sur la place publique ; il y a aussi la détresse d'une épouse et l'espérance d'une mère. Reconnaître, car reconnaissons que ni le droit ni la médecine ne nous offrent des réponses indiscutables. L'institution médicale est divisée. Quant à l'institution judiciaire, l'arrêt rendu hier soir par la cour d'appel de Paris démontre que, sur le plan du droit également, des interrogations demeurent. Alors, qui croire ? Que croire ? Il n'y a pas, mes chers collègues, de certitudes. Qui sait ici, dans cet hémicycle, ce que veut Vincent Lambert ? Qui pourrait affirmer savoir ce que les médecins eux-mêmes ne savent pas ? Ayons la force d'esprit et de coeur d'admettre que nous ne savons pas. Peut-être devrions-nous nous interroger avec humilité sur deux questions fondamentales que je vous pose, madame la ministre ? D'abord, jusqu'où pouvons-nous considérer qu'une vie ne vaut plus la peine d'être vécue ? Par ailleurs, l'incertitude, le doute et les décisions parfois contradictoires dans cette terrible affaire font craindre à beaucoup de Français le risque d'une dérive préjudiciable aux plus fragiles, une sorte d'insécurité éthique.

santé. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bernard Fournier, je crois pouvoir le dire, comme beaucoup de Français, nous sommes nombreux ici à être bouleversés par cette situation, par ce drame familial, qui touche à l'intime de chacun d'entre nous. Vous le savez, l'État français a toujours été soucieux de s'assurer que l'application de la procédure d'arrêt de traitement en cas d'obstination déraisonnable respectait le cadre de la loi Claeys-Leonetti, votée en 2016. Hier soir, la cour d'appel de Paris a accepté la requête des parents de Vincent Lambert et a ordonné la reprise des traitements, afin de respecter les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. L'équipe médicale en charge de Vincent Lambert appliquera ces mesures provisoires. Je n'en dirai pas davantage sur ce cas particulier. Aujourd'hui, encore plus que jamais, nous devons respecter l'intimité et la douleur de la famille et des proches de Vincent Lambert. La seule leçon que nous pouvons retenir de cette situation, c'est que chacun remplisse ses directives anticipées. Chaque personne majeure peut, depuis la loi Claeys-Leonetti de 2016, rédiger par avance une déclaration pour préciser ses volontés en fin de vie. Chacun peut inscrire son refus ou sa volonté de poursuivre, de limiter ou d'arrêter les traitements ou les actes médicaux. Les consignes données dans les directives anticipées permettent aux équipes médicales de prendre en charge les patients en respectant leur propre volonté.

des mesures sur la régulation des réseaux sociaux. Celles-ci font suite à une mission effectuée auprès de Facebook. Le rapport publié ce mois-ci a été salué par l'entreprise comme « un modèle pour la régulation des contenus en Europe Ces mesures prônent une simple corégulation de ces plateformes. Surprenant, très surprenant, au moment où des voix s'élèvent des deux côtés de l'Atlantique pour dire l'impossibilité d'une ou d'une corégulation de cette société. C'est le cas de la sénatrice Elizabeth Warren ou encore de Chris Hughes, un des cofondateurs de Facebook, qui va lui-même jusqu'à réclamer son démantèlement. Ce rapport évite soigneusement d'aborder la question du modèle économique de cette société.

très regrettable, si l'on considère les graves dérives éthiques, économiques et politiques dont s'est rendu coupable Facebook avec l'affaire Cambridge Analytica, affaire à laquelle a été lié un certain Steve Bannon. Il est illusoire de penser que la société peut remettre elle-même en cause son propre modèle basé sur toujours plus de données collectées, et donc toujours plus de gains. Mes questions sont simples. Compte tenu des enjeux pour la souveraineté de la France, quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre un terme à ces pratiques régulières de pantouflage, puis de rétropantouflage de notre haute administration, notamment avec les Gafam ? N'est-il pas temps de sortir de la complaisance pour prendre des mesures de régulation réellement contraignantes sur le coeur même de l'activité de ces sociétés, comme annoncent vouloir le faire, d'ailleurs, nos voisins allemands, depuis toujours beaucoup plus lucides et exigeants que nous sur le sujet ?

Inédits, car la complexité technologique des outils de ces acteurs est sans cesse croissante. Pour autant, et vous l'avez rappelé, les questions posées par ces acteurs sont très concrètes et ont impact sur nos concitoyens dans leur quotidien. Je suis persuadé d'une chose, madame la présidente, c'est que l'émergence de ces acteurs impose une obligation de résultat aux démocraties pour une raison simple simple : si les seuls États qui savent efficacement réguler les grands acteurs de l'internet- réseaux sociaux et plateformes -sont les pouvoirs autoritaires, alors, nos citoyens se tourneront vers des solutions autoritaires.

Nous devons donc en appeler à la responsabilité individuelle. Il n'est pas possible aujourd'hui que l'on puisse impunément insulter, injurier sur internet, sans que la justice vienne vous demander des comptes. Cela nécessite de poser des règles claires, et l'État

l'influent site d'actualité économique En tout état de cause, fallait-il absolument dérouler le tapis rouge à Mark Zuckerberg, qui s'est, je le rappelle, parjuré devant le Congrès

En Autriche, le vice-chancelier a dû démissionner à la suite d'une collusion avec un État étranger qui tente régulièrement de déstabiliser nos démocraties, notamment internet, ce qui n'est pas sans lien avec la question précédente. Il est reproché au vice-chancelier autrichien non seulement de s'être aventuré à des promesses, mais aussi de mettre en péril la confidentialité des informations dont ses services ont pu avoir connaissance. l'Autriche est écartée de certaines réunions et de certaines informations, qui sont communiquées, notamment, par le gouvernement allemand. Cette affaire est donc profonde et grave. Elle touche à la souveraineté et à l'indépendance de l'Europe. Les nationalistes se font les ennemis de l'intérêt national, qu'ils liquident au profit de leurs intérêts personnels et au profit de puissances étrangères. Ma question est double, À court terme, quelle est la position de notre pays face à la crise de la coalition autrichienne, notamment au regard du fonctionnement des institutions européennes, en particulier le Conseil ? Par Par ailleurs, l'influence d'États étrangers dans le déroulement régulier d'élections, et plus largement dans la vie politique, pose question. Le Parlement sera-t-il informé

et des affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Julien Bargeton, les citoyens européens sont libres et souverains, et ils entendent bien le rester. Les États européens sont libres et souverains, et ils entendent bien le rester. Cela paraît une évidence, ici dans cet hémicycle, mais les événements de ce week-end, effectivement, sont préoccupants. Préoccupants, parce que l'on voit les ingérences

Un certain nombre de mesures ont été prises : dispositions législatives visant à prohiber le financement par des établissements bancaires en dehors de l'Union européenne mise en place d'un réseau d'alerte européen pour s'informer des attaques détectées. Il est temps d'aller plus loin au niveau de l'Union. Le Président de la République a ainsi souhaité la création d'une véritable agence de protection

des peuples européens, alors, n'en déplaise à Marine Le Pen, une Europe européenne ne fait pas de génuflexions devant M. Bannon ; une Europe européenne ne se compromet pas, comme ses alliés autrichiens au Parlement européen ; une Europe européenne est unie, démocratique et libre

Avec 115 cas environ par an, notre pays était considéré jusque-là comme relativement stable, mais le nombre de cas augmente. La Nouvelle-Aquitaine est la région de France la plus touchée par ce phénomène. Après la Charente et la Dordogne, le département de la Gironde découvre quelques cas. Fabienne est maire de son village, mais elle est aussi éleveuse dans le Libournais. Elle est à la tête d'une petite exploitation et elle vit dans l'angoisse. Elle a dû faire face à l'abattage d'une vache. Une vache, me direz-vous, ce n'est rien, mais pour Fabienne, c'est tout ! D'autant que sa vache a été sacrifiée pour rien, parce qu'en fait elle n'était pas tuberculeuse. Elle était une « fausse positive ». Eh oui, la technique de nos tests date d'une cinquantaine d'années, et elle n'est pas totalement fiable. Monsieur le ministre, il nous faut investir très vite la question de l'actualisation des moyens de dépistage de la tuberculose bovine et de leur fiabilité.

recommande d'ailleurs d'effectuer des prélèvements sur un échantillonnage représentatif de cet animal autour des zones d'abattage. Nous attendons avec impatience les décisions sur le terrain en la matière.

Monsieur le ministre, alors que la filière est confrontée à une baisse de 12 % de la consommation de viande sur ces dix dernières années et qu'elle doit faire face aux dérives sans précédent de l'intolérance animaliste, quels moyens

de tuberculose bovine. Elle l'est depuis 2001, et il n'y a aucune raison qu'elle ne le reste pas. En tout cas, tous les services travaillent entre eux- services publics et services privés, ainsi que fédérations de chasse,

de trop ! -qui ont été mis en évidence sur le territoire national, soit une augmentation de près de 30

Je souhaiterais à mon tour interpeller Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Madame la ministre, en fin de semaine dernière, près de 50 000 lycéens ont fait les frais d'un bug de Parcoursup. À la mise en place de ce nouveau dispositif, nombreuses étaient les personnes à s'émouvoir de l'impact psychologique de l'attente des réponses et de la vérification des classements. Mais qui aurait pu prévoir un tel ascenseur émotionnel pour ces jeunes gens à un mois du début des épreuves du baccalauréat ? Comment en est-on arrivé là, moins de deux ans après le fiasco d'Admission post-bac, APB ? Les témoignages de lycéens déçus et de familles inquiètes affluent. En filigrane se dessine de nouveau la grande interrogation à propos des algorithmes et du manque de transparence de la plateforme.

Nous sommes nombreux à nous demander si les formations n'ont pas été sciemment encouragées à gonfler excessivement leur taux de surréservation pour raccourcir les délais d'attente pour les candidats et accélérer la fameuse convergence.

comme les responsables de ces formations ont réagi immédiatement de façon à ce que l'ensemble des 900 000 candidats puissent, avec quelques heures de retard,

les responsables de formation, les professeurs principaux et les proviseurs des lycées qui accueillent ces jeunes. Je voudrais les saluer aujourd'hui.

ou de classes préparatoires à 30 places qui ont appelé plus de 600 candidats, à cause d'une interversion du chiffre d'appel et du chiffre de la liste d'attente.

vous avez annoncé plusieurs mesures concernant le tourisme, et notamment un assouplissement des mesures de détaxe pour les touristes étrangers hors Union européenne. Nous ne pouvons que saluer cette initiative, qui devrait soutenir notre balance des paiements et la consommation. En effet, la France demeure la première destination touristique au monde en nombre de touristes, mais pas en recettes, où nous sommes derrière l'Espagne, un concurrent direct. Tout l'enjeu est ici de rétrécir l'avantage concurrentiel de nos voisins sur les conditions de détaxe. Aussi l'optimisation du mécanisme de la détaxe va-t-elle permettre une augmentation des sommes dépensées par les touristes. En 2018, près de 56,2 milliards d'euros ont été dépensés en France par les touristes étrangers. Monsieur le secrétaire d'État, quels sont les objectifs pour les prochaines années en matière de dépenses des touristes étrangers en France ? Par ailleurs, plus de 100 000 emplois ne sont pas pourvus dans le secteur touristique, et notamment dans l'hôtellerie-restauration. Vous avez annoncé plusieurs mesures, telles que la création d'un comité de filière pour le tourisme, la mise en place d'une plateforme numérique, ou l'instauration d'un contrat liant une douzaine de branches relevant du secteur du tourisme. Pouvez-vous nous préciser le calendrier de ces mesures et les objectifs du Gouvernement en matière d'emploi ? Comme vous l'avez précisé à plusieurs reprises, les problèmes de recrutement du secteur touristique sont essentiellement dus aux conditions de travail et de rémunération des emplois offerts. Des avancées significatives sont-elles attendues concernant l'attractivité de ces emplois ? La parole

France. Le comité interministériel du tourisme, réuni sous l'autorité du Premier ministre vendredi dernier, a pris un certain nombre de mesures afin d'atteindre des objectifs ambitieux,

des mesures très concrètes ont été prises, pour favoriser l'achat. Il faut avoir en tête que les touristes dépensent seulement 20 % de leur budget

Cette ambition touristique se décline également en matière de ressources humaines. Vous avez raison, nous ne pouvons pas nous résoudre à voir 100 000 emplois non pourvus dans ce secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les professionnels du tourisme se sont emparés du sujet

Manifestement, ni la honte d'une condamnation pénale ni la peine prononcée ne l'auront amené à réfléchir. En effet, le rappeur, homme libre, comme il aime à se présenter lui-même, vient de réitérer son propos dans son nouveau clip aux paroles sans ambiguïté : « Je baise la France ; je brûle la France jusqu'à l'agonie ». Tel est le refrain lancinant de ce qu'il présente comme une oeuvre de l'esprit. Au-delà des propos tenus, les images laissent peu de place à l'interprétation. Dans ce clip, à large diffusion, on voit l'auteur, après sa déambulation en berline, clamer sa haine de la France, et procéder avec méthode à la strangulation d'une jeune femme à terre, le tout suivi d'un ralenti complaisant laissant apparaître son rictus de satisfaction devant son crime. Amené à s'expliquer sur ces propos et ces images, l'auteur invoque tour à tour la faute des médias et de la mentalité française, qui, selon lui, refuserait « d'ouvrir le sujet épineux de l'esclavagisme de la France ». Monsieur le secrétaire d'État, on ne saurait en pareil cas s'abriter derrière la liberté de création ou la liberté d'expression pour tout justifier. Les limites ont, me semble-t-il, été largement été outrepassées.

L'insulte et la haine ne sont pas de l'art. L'insulte et la haine ne vont pas dans le sens du « vivre ensemble » auquel nous appelons tous dans notre démocratie française. Mais surtout, l'insulte et la haine tombent sous le coup de la loi pénale. C'est en ce sens que Christophe Castaner a, dès dimanche, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, saisi le procureur de la République de Paris, qui a immédiatement

Vous reportiez alors l'application des recommandations de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, à savoir l'augmentation des tarifs. En juin prochain, vous allez valider les nouveaux tarifs, soit une augmentation considérable de 5,9 %, majorée de 1 % supplémentaire en août. Cela signifie une augmentation de 85 euros par an pour un ménage qui se chauffe à l'électricité, une hausse que la récente augmentation du chèque énergie, d'un montant de 50 euros, ne permettra pas de compenser. Ces hausses de tarif sont très largement contestées. Elles le sont directement par le Médiateur national de l'énergie et par les associations de défense des consommateurs, qui alertent sur la baisse du pouvoir d'achat subséquente. indirectement par l'Autorité de la concurrence, qui s'est élevée contre les changements de méthode et d'analyse de marché adoptés par la Commission de régulation de l'énergie et responsables de cette forte hausse des tarifs. Ces augmentations sont le fruit d'un mécanisme imposé pour favoriser la concurrence, au détriment, bien sûr, des consommateurs. Or la précarité énergétique est une triste réalité. Elle touche 3,3 millions de ménages en France, soit 6,7 millions de personnes qui restreignent leur utilisation de chauffage, ont froid dans leur logement, vivent dans une seule pièce l'hiver et s'endettent

Par ailleurs, vous avez parlé de modifier le mode de calcul des tarifs de l'électricité sans rien préciser de vos intentions. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le pouvoir d'achat, c'est le travail. La philosophie de ce gouvernement et de cette majorité, c'est de passer par le travail et par l'emploi pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et vous devriez vous réjouir

Le Président de la République vient également d'annoncer une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu pour tous ceux qui travaillent. Vous le voyez, au-delà du sujet de l'énergie, la question clé pour nos compatriotes, pour tous ceux qui vont travailler, qui ont un emploi, qui sont salariés, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail. Eh bien, c'est l'honneur de cette majorité que de permettre à tous ceux qui travaillent de vivre dignement de leur emploi ! C'est notre philosophie, c'est notre politique et ce sont nos résultats

Cette situation amène quatre sujets dangereux pour notre vision régalienne et protectrice de la santé. Primo, la plateforme permet la prise rapide de rendez-vous de consultation à toute heure du jour ou de la nuit. Cela plaît, mais est-ce souhaitable ? En effet, une réponse immédiate à un besoin de santé oublie la prévention, la prise en compte des habitudes de vie, l'histoire du patient, l'éducation thérapeutique.

Tertio, la plateforme contractualise avec des cliniques, établissements de santé, hôpitaux publics, dont les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'AP-HP. Quand un patient se rend sur le site de l'AP-HP, par exemple, pour prendre rendez-vous, il doit créer un compte Doctolib. Ainsi, les patients de l'AP-HP doivent s'inscrire sur un site privé, alors que l'hôpital public, faut-il le rappeler, est financé par l'argent public ? Il y a là, me semble-t-il, un problème éthique grave. Enfin, cette alliance entre cliniques, hôpitaux, professionnels de santé et Doctolib crée un risque majeur pour la protection des données de santé. En effet, la plateforme collecte les données personnelles des patients, le nom de leur médecin, le motif de consultation ou d'examen complémentaire, mais aussi les comptes rendus des téléconsultations.

Madame la ministre, il y a urgence ! Avant qu'il ne soit trop tard, quelles mesures comptez-vous prendre pour sécuriser les patients et les pratiques médicales face à cette évolution et au risque d'ubérisation de la santé ? La parole

Vous prenez l'exemple de la plateforme de rendez-vous en ligne. En France, vous le savez, les données de santé sont très encadrées grâce au règlement général européen sur la protection des données, le RGPD. Les données de santé sont encore davantage encadrées, puisque chaque société qui en récolte est chargée de les chiffrer et de les stocker chez un hébergeur agréé. Les données personnelles de santé des utilisateurs sont ainsi validées par des prestataires ayant reçu un agrément certifié « hébergeur de données de santé » et leur exploitation est très surveillée. Les plateformes auxquelles vous faites référence respectent l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires françaises et européennes relatives à la protection des données personnelles. Madame la sénatrice, je suis également très attachée à la protection des données. Je voudrais prendre pour exemple ce que nous avons fait dans le projet de loi Santé que vous serez amenés à examiner dans une semaine. L'article 11 de ce texte, qui est dédié au Health Data Hub, vise justement à parvenir à un équilibre entre les usages innovants et efficaces des données de santé, en vue d'améliorer nos connaissances et la protection de la vie privée. Cet équilibre a d'ailleurs été salué par le Conseil d'État. Il a considéré que le projet de loi ne méconnaît aucune exigence de valeur constitutionnelle ou conventionnelle, dès lors que le système national des données de santé apporte des garanties suffisantes pour l'utilisation des données auxquelles il donne accès. vous aurez tout le loisir de le vérifier lors des discussions parlementaires, nous serons extrêmement vigilants à ce qu'aucun Français ne soit inquiété quant à l'utilisation de ses données de santé. C'est ce que nous devons à nos concitoyens. La parole

la tyrannie subie par certaines femmes avec la liberté dont disposent d'autres femmes, les agents du service public avec les maires bénévoles- sans aucune arrière-pensée ... Et on finira par confondre Mme Ibn Ziaten avec des salafistes et lui empêcher l'accès aux établissements

Il a été indiqué que mon collègue Franck Menonville et moi-même, pour le groupe Les Indépendants, n'avions pas pris part au vote. Or nous souhaitions voter pour

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés

nous examinons aujourd'hui en séance publique le projet de loi sur la taxation des géants du numérique et sur la modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. avoir suivi attentivement vos débats en commission, j'ai vu émerger deux grandes inquiétudes auxquelles je voudrais répondre, car je n'aime pas voir des sénateurs inquiets

et c'est l'engagement qu'il a pris au cours de sa campagne présidentielle. Cet engagement sera tenu non par obstination, mais tout simplement parce qu'il donne des résultats. La seule manière de consolider notre économie et la compétitivité de nos entreprises tout en garantissant prospérité et emploi à nos compatriotes, c'est de maintenir une politique de l'offre,

le taux de l'impôt sur les sociétés sera de 25 % pour toutes les entreprises françaises, sans exception, en 2022. C'est l'un des enjeux majeurs de compétitivité pour notre économie et c'est l'une des conditions du rétablissement de notre attractivité. Si nous attractivité. Si nous entrons enfin pour la première fois dans le top 5 des nations les plus attractives de la planète, c'est précisément parce que nous avons une politique fiscale attractive et que nous tenons nos engagements : un impôt sur les sociétés à 25 en 2022 pour toutes les entreprises, même les plus grandes d'entre elles. Certains nous ont reproché, en décalant la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés,

précisément pour avoir un coût du travail compétitif par rapport à nos grands concurrents européens. C'est bien l'intégralité du CICE qui sera transformée en allégement de charges, ce qui évitera les décalages de trésorerie pour les entreprises et nous permettra d'avoir un coût du travail aussi compétitif que celui de nos voisins allemands. Le choix de la suppression de l'impôt sur la fortune, l'ISF, a été maintenu et Dieu sait qu'il a pu être contesté ! La création d'un prélèvement forfaitaire unique pour les revenus du capital à 30 % a été maintenue. Tous les éléments fondamentaux de la politique de l'offre- taux de 25 % pour toutes les entreprises, l'allégement de la fiscalité sur le capital, la transformation du CICE en allégement de charges -ont donc été maintenus par le Président de la République, confirmant le cap d'une politique de l'offre pour la nation française.

Votre seconde inquiétude concernait la taxation même des géants du numérique, qui est au coeur de nos discussions aujourd'hui. Vous avez mentionné plusieurs éléments de préoccupation auxquels je voudrais répondre.

les géants du numérique, qu'ils soient américains, européens ou chinois, paient quatorze points d'impôt en moins que nos grandes entreprises, nos PME, nos TPE ou nos commerces. Ce n'est pas normal ! C'est inacceptable et je ne m'y résignerai jamais.

la Commission européenne à déposer, en janvier 2018, une proposition de taxation des géants du numérique. Celle-ci reposait sur le chiffre d'affaires,

Dans les mois qui ont suivi, nous avons essayé d'entraîner l'intégralité de nos partenaires européens, puisque les décisions fiscales se prennent à l'unanimité,

j'ai proposé au Président de la République et au Premier ministre que, comme l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Espagne, nous prenions une disposition nationale,

et sur lesquels le Conseil d'État nourrissait des doutes. Il est vrai que proposer des services financiers sur internet ne crée pas nécessairement de la valeur par effet de réseau et donc n'entre pas dans le champ de la taxe. Pour ces raisons, nous estimons

Troisième élément d'inquiétude : la taxe nationale serait dangereuse pour la compétitivité de nos entreprises. Je tiens simplement à indiquer que nous avons défini le champ le plus responsable possible et, surtout, que nous avons ciblé les entreprises dont le chiffre d'affaires numérique,

Cette taxation du numérique est la première brique de la construction d'une taxation internationale conforme à cet objectif : il n'est pas acceptable que des géants du numérique utilisent les données des Français et ne paient pas au Trésor public français leur juste part d'impôts.

Vous l'avez rappelé, il est apparu clairement, en décembre dernier, que la solution temporaire proposée par la Commission ne pouvait être acceptée- je ne reviens pas sur le problème de la règle de l'unanimité ; le Gouvernement a donc proposé de transcrire cette proposition européenne dans notre droit national.

de lever l'impôt, remettant ainsi en cause l'un des aspects essentiels de la fiscalité : son caractère national. Ces défis, le Sénat les connaît. Beaucoup de nos collègues ont travaillé sur ces questions, particulièrement au sein de notre commission des finances. Je salue ici le travail fait dans le passé et le travail d'aujourd'hui. Les amendements qui ont été présentés par le rapporteur en sont une illustration fidèle. À titre d'exemple, en 2012, le rapport d'information de Philippe Marini sur la fiscalité numérique concluait que les entreprises du numérique étaient, en Europe, assujetties à un taux moyen de 9 % pour l'impôt sur les sociétés, alors que ce taux s'élevait à 23 % pour les entreprises dites traditionnelles du secteur physique.

qui est menacé, alors que chaque atteinte aux principes fondateurs de notre République est vécue comme une injustice insupportable par nos concitoyens. L'économie numérique est l'économie de demain, ne pas s'intéresser à la taxation du numérique et attendre les autres pays serait une véritable capitulation. Il revient aux responsables politiques de répondre à ces injustices et c'est ce que vous avez fait, monsieur le ministre, avec le gouvernement auquel vous appartenez. Vous présentez au Parlement un texte de justice fiscale, mais aussi d'efficacité. Justice, face au différentiel de quatorze points entre les entreprises numériques et les entreprises traditionnelles dans le paiement de l'impôt ; efficacité,

Plus il y a de recherches, plus la plateforme est valorisée et plus elle est monétisable par des annonceurs. Cet effet de réseau se fait sans présence physique et permet d'éviter l'impôt en France

et c'est ce que vous faites, monsieur le ministre. Cette taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires numérique réalisé en France ne touchera que les plus grandes entreprises du numérique grâce au double seuil cumulatif. Ne seront assujettis que les secteurs créant le plus de valeur : la publicité ciblée en ligne, la vente de données à des fins publicitaires et la mise en relation des internautes par les plateformes. Cette taxe sur les services

outre, il ne répond pas à la possibilité dont disposent ces entreprises de déplacer leur résultat dans des pays à faible fiscalité ou de délocaliser les bénéfices dans des paradis fiscaux. Si nous décidons de taxer ces entreprises qui ne paient pas leur juste part d'impôt, c'est parce que les règles de l'impôt ne sont plus adaptées à l'économie. Ainsi, et en suivant le droit, le 12 juillet 2017 le tribunal administratif de Paris a jugé que Google Irlande ne disposait d'aucun établissement stable en France, parce que Google France ne pouvait engager juridiquement la société et a ainsi annulé le redressement fiscal de plus de 1 milliard d'euros infligé à Google par le fisc français. Dès lors que le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés françaises exempte les bénéfices réalisés par une société française lorsqu'ils le sont au moyen d'une entreprise exploitée à l'étranger, il est difficile de ne pas accepter la réciproque. Ces règles nouvelles devront émerger d'un cadre multilatéral. Celui-ci existe : c'est l'OCDE, laquelle, après avoir défini un plan d'action en juillet 2013 2013 contre l'érosion des bases en matière de fiscalité des entreprises, a lancé très récemment un programme de travail pour trouver une solution technique. Plusieurs modèles s'opposent : l'un fondé sur la « participation de l'utilisateur

Ces modèles reposent sur des conceptions opposées de l'économie numérisée et de la manière dont elle doit être fiscalisée. Dans quelle mesure la valeur provient-elle de la participation de l'utilisateur par l'effet de réseau que j'ai évoqué et relativement aux aux biens de commercialisation ? Les pays membres de l'OCDE devront trancher d'ici deux ans. En attendant, la France doit appliquer une mesure temporaire de justice entre les entreprises traditionnelles et celles du numérique. En commission des finances, nous avons complété le texte par des dispositions utiles, comme l'application de la règle de détermination du coefficient de présence numérique pour l'année 2019 à l'assujettissement et non à la seule liquidation. Notre groupe votera ce projet

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les acronymes sont parfois trompeurs. Ainsi, nous devrions discuter de la mise en place d'une taxe visant les Gafa,

La proposition de taxation du numérique découle de la même logique : l'affichage plutôt qu'une fiscalisation efficace. De fait, les grandes firmes multinationales sont épargnées, au détriment de leur contribution à la solidarité nationale. Mes chers collègues, si le principe d'une taxe sur les services et activités numériques est juste et nécessaire, ce projet de loi ne permettra pas, en l'état, d'atteindre les objectifs ambitieux auxquels il doit tendre. en effet, est beaucoup trop restreinte, alors que l'économie numérique s'apparente à une nouvelle révolution industrielle : les modes de production, d'échanges et d'implantation des firmes se transforment. En France, trois entreprises sur cinq sont passées au et 5,5 % du produit intérieur brut découlent directement du numérique. Surtout, le distinguo entre numérique, services et économie productive est désormais largement dépassé dans la réalité des grandes firmes françaises et européennes. Votre projet, monsieur le ministre, étroitement centré sur les interfaces numériques permettant aux utilisateurs d'entrer en contact entre eux et d'interagir directement, laissera de côté de grandes firmes multinationales très actives dans la sphère numérique, qui échappent déjà largement à l'impôt. À titre d'exemple, Netflix, PayPal ou encore Apple n'entrent pas dans le champ de ce que vous proposez ! Vous vous Vous vous targuez de modernité, mais, en réalité, vous êtes en retard sur l'évolution des marchés et de l'économie ... Ainsi, au-delà de l'assiette, les seuils retenus sont bien trop élevés pour appréhender effectivement les acteurs du numérique dans leur diversité.

pourquoi un tel cadeau, alors qu'il était possible d'inscrire dans la loi l'impossibilité d'une telle déductibilité ? Pourquoi un tel soutien, alors que, en moyenne, les grands groupes du numérique bénéficient d'un écart d'imposition de près de quatorze points par rapport aux entreprises suivant un modèle traditionnel ?

Alors que des États membres importants comme l'Espagne, l'Autriche et l'Italie ont prévu des dispositifs similaires, on sent un manque de motivation, qui nous amène à nous interroger sur les ambitions réelles du Gouvernement.

À cet égard, la taxe sur les services numériques qui nous est proposée va dans le bon sens, mais reste très insuffisante ; on ne peut manquer de s'interroger, à la suite de la commission elle-même, sur sa portée réelle. Ensuite, ce projet de loi s'inscrit dans le financement des mesures annoncées en décembre dernier par le Président de la République pour faire face à la colère sociale. Seulement, sur ce point, le compte n'y est pas ... De fait, nous sommes

Nous ne pouvons que constater l'échec de la France à mettre en oeuvre, avec nos partenaires européens, ce projet d'établissement stable numérique permettant de taxer les bénéfices

Nous trouvons juste que les bénéfices de ces grandes entreprises soient imposés davantage, afin de participer aux mesures sociales revendiquées par nos concitoyens. Nous savons que le taux d'impôt sur les sociétés ne représente qu'une partie de l'équation, mais il en est la partie la plus visible.

pour présenter cette suspension de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Disons aussi qu'une entreprise multinationale investit dans un État pour la qualité de la formation de ses citoyens et celle de ses infrastructures, qui supposent des ressources fiscales et une juste répartition

représente un véritable défi pour les systèmes fiscaux actuels, dont les fondements remontent à l'après-guerre. Alors que le prélèvement de l'impôt, en France, repose sur le principe de territorialité, selon lequel la localisation des biens et activités permet de déterminer les contributions obligatoires, les sociétés du numérique peuvent opérer auprès d'utilisateurs situés en France sans être nécessairement implantées dans l'Hexagone ou, plus précisément, sans y avoir d'établissement stable. Si les problèmes liés à l'optimisation fiscale par le biais d'implantations dans des pays à fiscalité plus avantageuse et par le moyen des prix de transfert intragroupe le défi posé par l'économie numérique est encore plus grand, si l'on en juge par les montants d'impôt assez faibles payés par ces grandes entreprises au regard de la valeur créée. La définition des activités taxables est particulièrement importante et complexe. Le Gouvernement a choisi d'y inclure le ciblage publicitaire et la mise en relation des utilisateurs, mais non la vente en ligne. Par ailleurs, plusieurs types de services proposés par les plateformes ne sont pas taxables : la fourniture de contenus de type YouTube ou Dailymotion et les services de communication comme Skype, ou encore les services de paiement. les services de paiement. La directive européenne sur les services de paiement, dans sa deuxième version, a été transposée l'an dernier. D'autres activités, comme le conseil en financement participatif, sont également exclues du champ de la taxe. L'idée générale reste d'appliquer une taxe aux activités qui se rapportent à une forme de travail gratuit des utilisateurs, créateur de valeur. Diverses tentatives ont été faites

Finalement, le gouvernement français, comme d'autres gouvernements européens, a décidé de légiférer au niveau national. À ce jour, l'Italie semble avoir le projet le plus abouti, avec une censée entrer en vigueur en juin prochain. Dans le présent projet de loi, l'assiette choisie, une estimation du chiffre d'affaires réalisé en France à partir d'un pourcentage représentatif du chiffre d'affaires mondial, vise à reterritorialiser le chiffre d'affaires. de la valeur ajoutée, qui aurait été plus satisfaisante, ni du bénéfice, dont la territorialisation est beaucoup plus difficile à appréhender. Cette approche repose sur l'hypothèse qu'il existe une proportionnalité entre le nombre de transactions et les sommes encaissées, dans l'attente de la reconnaissance d'un établissement stable virtuel. La démarche de la France n'est pas originale en soi. Le débat sur la taxation des Gafa existe depuis plusieurs années, et d'autres pays européens poursuivent des projets similaires, bien qu'une différence se remarque entre les pays du nord de l'Europe, peu enclins à instaurer cette taxe, et les pays latins, plus avancés dans cette voie. Quoi qu'il en soit, l'objectif est avant tout d'accélérer une mise en oeuvre collective de cette taxation, malgré un contexte mondial marqué par des tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine. En Europe, on espère un redémarrage du projet de directive, peut-être après les élections de dimanche prochain. On ne peut pas reprocher aux Français et à la France, et plus largement aux Européens, de vouloir jouer un rôle précurseur dans la réalisation d'une plus grande équité fiscale, alors qu'on demande par ailleurs plus de rigueur budgétaire. Plus globalement, les négociations doivent être poursuivies dans le cadre de l'OCDE, ce qui justifie, à mon sens, la modification proposée par le Sénat en ce qui concerne le caractère temporaire de ce dispositif.

Il est vrai que la réponse devrait être apportée à l'échelle mondiale ; mais nous savons que, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour y parvenir. Plusieurs pays, et non des moindres, ne sont

qu'il ne faut rien changer, comme nous l'entendons parfois ? Je ne le crois pas. Ni la complexité de la mise en place, ni les positions contraires d'autres pays, ni même la prise de risque ne doivent nous conduire à renoncer !

donne. Par ailleurs, c'est une question d'équité fiscale, un sujet sur lequel nos concitoyens sont mobilisés et réclament, à juste titre, davantage de justice. Au reste, l'équité fiscale se joue aussi entre les entreprises qui paient déjà leurs impôts en France et celles, les géants du numérique, qui profitent du lucratif marché français sans participer au bon niveau à l'effort collectif. Il n'est pas tenable, sous le seul prétexte de la complexité ou de l'impossibilité d'un accord européen ou mondial, de continuer à taxer nos entreprises traditionnelles, nos PME, nos artisans et nos commerçants sans traiter le cas des géants du numérique ! Enfin, on ne peut pas, d'un côté, se fixer comme objectif majeur de réduire notre déficit et, de l'autre, se priver de la recette fiscale légitimement due par les géants du numérique. En adoptant cette taxe, la France adresserait à l'ensemble de ses voisins un signal fort, donnant par la même occasion une impulsion qui pourrait s'avérer décisive dans l'adaptation du cadre fiscal international au déploiement de l'économie numérique. Alors, oui, malgré les difficultés, la France doit s'engager sans attendre sur la voie de la taxation des grandes entreprises du numérique. Pour ce faire, monsieur le ministre, vous nous proposez d'instaurer une taxe sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros au titre des services fournis au niveau mondial et à 25 millions d'euros au titre des services fournis en France. Cette taxe représentera 3 % sur les produits bruts tirés des services de ciblage publicitaire, de la transmission de données personnelles et de l'activité des places de marché du commerce en ligne. Certes, comme plusieurs orateurs l'ont souligné, l'assiette retenue n'est pas la solution idéale. Taxer le chiffre d'affaires, c'est taxer sans distinction l'entreprise en pleine croissance qui n'enregistre pas ou peu de résultats et celle dont les résultats sont élevés. La taxation des bénéfices eût été préférable ; mais, nous le savons, elle nécessiterait la renégociation de conventions fiscales bilatérales.

et à limiter à trois années sa première mise en application- nous en reparlerons dans la discussion des articles. Mes chers collègues, face aux géants du numérique, qui se jouent des règles fiscales traditionnelles,

même s'il ne s'agit que d'un premier pas, avec une recette estimée à 400 millions d'euros en 2019, et qu'une solution internationale doit être trouvée. J'en viens à l'article 2 du projet de loi, qui prévoit de déroger à la trajectoire de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés pour les plus grandes entreprises, celles réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, et seulement pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 500 000 euros. Il leur serait appliqué, pour la seule année 2019, le taux de 2018, soit 33,33 %. J'entends l'argument selon lequel, pour donner de la visibilité aux acteurs économiques, on ne devrait pas changer les règles du jeu en cours de route. Évidemment, nous partageons tous cet objectif. Mais nous pouvons aussi considérer que nous avons une exigence de responsabilité au regard de notre déficit public, que nous souhaitons tous diminuer

constitue ainsi un levier utile, parmi d'autres, pour compenser la dépense substantielle que le Gouvernement et le Parlement ont décidée en faveur du pouvoir d'achat des Français.

nous examinons cet après-midi le projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.

Cette pression est d'autant plus inacceptable que certaines sociétés- de même que certains particuliers, mais ce n'est pas le sujet de cet après-midi -tentent de contourner l'impôt en pratiquant ce qu'on appelle l'évitement fiscal. Or, aujourd'hui,

nous voulons, avec cette taxation des géants du numérique, inventer la fiscalité du XXI siècle » ; vous venez de rappeler cette volonté. Cela dit, plus prosaïquement, ce projet de loi vise surtout à dégager des économies pour financer, en partie, les mesures de pouvoir d'achat adoptées en décembre dernier, au plus fort du mouvement des « gilets jaunes Vous l'admettiez vous-même le 6 mars : cette taxe « est une question d'efficacité pour nos finances publiques ». Les mesures de pouvoir d'achat adoptées au travers de deux textes représentent respectivement 3,7 milliards et 7,3 milliards d'euros, soit 11 milliards d'euros de nouvelles dépenses.

Nous sommes loin de l'équilibre ... Nous avons pris bonne note de la volonté du Gouvernement de réaliser 1,5 milliard d'euros d'économies sur le budget de l'État ; peut-être M. le ministre pourra-t-il nous apporter quelques informations à ce sujet, encore trop peu précisé et documenté. Les nouvelles mesures annoncées fin avril, à l'issue du grand débat national, vont doubler le montant de la facture, qui sera en réalité essentiellement financée par le déficit public, donc par la dette, les recettes nouvelles discutées ce soir n'ayant qu'un caractère temporaire. Aujourd'hui, seules les entreprises, notamment les champions français, sont mises à contribution pour payer la baisse de la fiscalité pesant sur les ménages. Cela passe tout d'abord par le report de la baisse de leur fiscalité : quel crédit sera donné, dans la suite du quinquennat, à la parole du Gouvernement ?

fiscales. Quant à la taxation des Gafa, il s'agit d'un serpent de mer. À l'instar de l'Union européenne ou de l'OCDE, le Sénat réfléchit depuis plusieurs années à la manière de mieux appréhender la capacité contributive des géants du numérique, face au développement rapide de ce secteur de l'économie. Les débats sont toujours très animés. très animés. Les règles internationales en vigueur permettent aux entreprises de rapatrier leurs impôts dans leur pays de production, alors qu'elles ne sont pas ou sont très peu taxées sur leurs lieux de consommation. C'est notamment pour cela qu'une société comme Google, pourtant très internationalisée, paierait, selon les données disponibles, 80 % de ses impôts aux États-Unis. Par ailleurs, ces sociétés profitent également des disparités des systèmes fiscaux européens pour faire de l'optimisation fiscale en transférant, de manière artificielle mais légale, l'essentiel de leur activité et de leurs bénéfices dans des pays où la fiscalité est plus accueillante, comme en Irlande ou au Luxembourg. Ces transferts sont facilités par le caractère immatériel des prestations commercialisées. La règle de l'unanimité qui prévaut en matière fiscale au sein de l'Union européenne, cela a été rappelé, n'a pas permis d'aboutir à un accord européen. Le projet de directive de mars 2018, qui prévoyait une taxe sur les services numériques à l'échelle européenne, a été rejeté par plusieurs États membres, notamment l'Irlande et les pays scandinaves. L'accord a été renvoyé à 2021. L'OCDE souhaite, pour sa part, trouver un accord international en 2020. 2020. À ces blocages politiques s'ajoute la difficulté d'établir un diagnostic réel de la fiscalité s'appliquant aujourd'hui aux Gafa. Selon le diagnostic établi par la Commission européenne, les géants du numérique paieraient en moyenne 14 points d'impôts de moins sur leurs bénéfices que les PME européennes le taux effectif moyen d'imposition des entreprises multinationales du secteur numérique serait en effet de 9,5 %, à comparer au taux moyen de 23,2 % pour les entreprises multinationales traditionnelles. Ce constat est contesté par l'Institut économique Molinari : selon cet organisme, les Gafa seraient en réalité imposés en moyenne à hauteur de 24 %, soit autant que les entreprises européennes. Les chiffres avancés par Bruxelles se fondent sur une étude du cabinet d'audit PwC et du laboratoire allemand de recherche en fiscalité ZEW. Cette étude a consisté à établir des simulations de la fiscalité des entreprises, sur le fondement des législations en vigueur les auteurs ont ainsi calculé que les entreprises numériques qui font beaucoup de recherche et développement, ou R&D, bénéficient d'une fiscalité très clémente de 12 % en France et de 9 % en Europe, contre 22 % aux États-Unis.

Les résultats de cet Institut montrent que les Gafa se sont acquittés de 24 % d'imposition sur leurs bénéfices mondiaux durant les cinq et dix dernières années. Cet Institut semble toutefois relativement isolé lorsqu'il écrit que le « niveau de fiscalité [des Gafa], loin d'être anormalement bas,

Par ailleurs, s'il peut être vrai que certaines entreprises étrangères font peu de bénéfices en France, ou n'en font pas, et, par conséquent, paient peu d'impôt sur les sociétés en France, elles s'acquittent pour autant de cette obligation ailleurs, conformément aux conventions fiscales négociées par la France. Mais oui. Notre pays profite aussi, en toute réciprocité, de ces conventions bilatérales, le versement de montants d'impôt sur les sociétés très importants acquittés par des groupes français ayant une activité en dehors du territoire français. Mettre en place une taxation spécifique contrebalançant les accords fiscaux que la France a signés pourrait donc être contre-productif, en provoquant des mesures de rétorsion de nos partenaires commerciaux, notamment des États-Unis. Les réactions américaines ont été très vives après l'annonce de la mise en place de cette taxe sur les services numériques par le gouvernement français, tant dans les milieux économiques que politiques, au Congrès notamment.

De surcroît, cette initiative française n'est pas sans poser de problèmes à nos propres entreprises. Faute d'avoir pu obtenir un accord à l'échelon européen, le Gouvernement propose une taxe nationale pour que les Gafa s'acquittent d'un impôt en France. Serait ainsi mise en place une fiscalité temporaire, en attendant une évolution des règles internationales de taxation, à l'échelon de l'OCDE, faute d'accord en Union européenne. L'assiette de cette taxe va toucher également des entreprises françaises du numérique en pleine croissance, alors même que la France manque encore d'entreprises Enfin, une taxe portant sur le chiffre d'affaires plutôt que sur les bénéfices frappera beaucoup plus fortement les entreprises qui ont des charges importantes, comme des locaux ou de nombreux À ce sujet, je ne peux manquer d'évoquer le risque juridique très sérieux, identifié par notre rapporteur, Albéric de Montgolfier, dont je tiens à souligner la qualité du travail sur un sujet qu'il connaît bien. Le seuil d'imposition fondé sur le chiffre d'affaires avantagera les entreprises situées au-dessous de ce seuil et pourrait entraîner une qualification d'aide d'État par la Cour de justice de Si la taxe était « retoquée » d'ici quelques années, la France devrait alors rembourser le montant des recettes perçues aux entreprises assujetties à la taxe, comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps. Le Gouvernement devrait sécuriser le dispositif en procédant à une notification auprès de la Commission européenne, comme l'y invite notre commission des finances. Au-delà du risque juridique, cette taxe mal préparée souffre également de difficultés techniques : la taxe sera calculée sur une base déclarative, qui, de manière pratique, sera quasiment impossible à vérifier pour l'administration fiscale. Aujourd'hui, les entreprises concernées ne sont pas encore dotées des outils informatiques permettant la consolidation de leur assiette taxable. Enfin, le rendement budgétaire de cette mesure pourrait être très inférieur aux recettes attendues.

Une taxe de 3 % rapporterait donc seulement 180 millions d'euros, et non 500 millions d'euros en moyenne, comme l'annonce le Gouvernement. Pour autant, malgré toutes ces réserves, le groupe Les Républicains soutiendra le principe de cette taxe, ... Très bien ! ... dans le seul espoir qu'elle permette d'accélérer les négociations au sein de l'OCDE. il est temps d'inventer cette « fiscalité du XXI siècle », une fiscalité qui n'ait pas seulement un objectif de rendement, aussi faible soit-il, mais également un objectif d'égalité. Les commerçants de nos centres-villes déplorent trop souvent l'inégalité entre leur régime fiscal et celui des géants du numérique ; ce projet de loi ne règle aucun des problèmes soulevés par le e-commerce. Le présent projet de loi contient une seconde mesure qui aura, elle aussi, un impact sur nos entreprises : son article 2 annule la baisse, prévue en 2019, de 33,3 % à 31 %, du taux de l'impôt sur les sociétés, pour l'ensemble des entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. L'engagement présidentiel d'Emmanuel Macron était une baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % en 2022, en passant par 31 % en 2019, conformément à la trajectoire définie dans la loi de finances pour 2018. En 2020, il était prévu En 2020, il était prévu que l'impôt sur les sociétés diminuerait à 28 %, mais, encore une fois, cela pourrait ne pas concerner toutes les entreprises. Monsieur le ministre, lors de la discussion du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré avez déclaré : « Je ne saurais prendre l'engagement que nous reprendrons, pour les seules entreprises réalisant plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, exactement la même trajectoire dans le PLF pour 2020 que dans le PLF pour 2018.

Les mesures de baisse de la fiscalité pesant sur les ménages ne doivent pas être compensées par des hausses de la fiscalité des entreprises. Notre niveau de fiscalité est le plus élevé du monde. Après le Danemark ! Nous devons globalement le faire diminuer. C'est à l'État de prendre ses responsabilités ; il ne faut plus attendre pour mettre en oeuvre de réelles économies, ce sont les seules mesures viables à long terme. Augmenter les impôts relève uniquement d'une vision de court terme ; les Français attendent un autre scénario que celui qui s'est déjà joué sous le quinquennat précédent.

Monsieur le ministre, vous les justifiez comme étant des mesures de rendement, de justice fiscale et de réponse aux décisions prises en décembre 2018 en faveur du pouvoir d'achat des ménages pour répondre à l'urgence sociale.

sûr ... Je ne reviens pas sur les propos de Rémi Féraud, que je partage. Au travers de l'article 2, vous rompez pour un an l'engagement pris par les différents gouvernements de baisse de l'impôt sur les sociétés.

À la question « La France s'apprête à taxer les Gafa. Est-ce une bonne idée ? », Jean-Baptiste Rudelle, PDG de Criteo, répondait dans un entretien au journal : « C'est la mauvaise réponse à deux bonnes questions. La première est une question générale qui concerne la taxation des multinationales. Sur un plan moral, il est normal que toutes les entreprises paient des impôts. [ ...] C'est un devoir, mais la réponse passe par une approche globale sur laquelle travaille l'OCDE. La seconde question est plus spécifiquement liée au monde du numérique. Les Gafa utilisent leur position dominante pour verrouiller une grosse partie de l'écosystème digital. Cela pose un vrai problème de souveraineté. » La fiscalité est devenue un sujet de préoccupation et les États n'ont pas su réagir rapidement à la mondialisation de l'économie et à la dérégulation financière ; ils sont plus rapides pour soutenir les banques, comme lors de la crise financière de 2007 et 2008 ... Nos systèmes fiscaux nationaux sont fondés sur une économie industrielle de production. Or l'introduction de l'internet et la numérisation de l'économie ont bouleversé un système fondé sur des conventions internationales, dont le modèle est issu de la crise de 1929. Ce modèle prévoit qu'une entreprise étrangère n'est taxable sur un territoire que lorsqu'elle y a un établissement stable, une présence physique. L'article 209 du code général des impôts correspond à ce principe : sont assujettis à l'impôt sur les sociétés les bénéfices tirés de l'exploitation d'une entreprise en France. Les décisions de justice récemment rendues à propos de Google démontrent, s'il en était besoin, les lacunes des conventions internationales et de notre droit fiscal. Votre proposition est une avancée, monsieur le ministre, même si nous regrettons cette politique des très petits pas. Nous ne pouvons que vous encourager dans la voie ouverte, déjà adopté, lors du débat sur la loi de finances pour 2019, un article destiné à avancer sur la voie de la taxation. Par ailleurs, en mai 2018, nous avions également soutenu la proposition de résolution européenne sur la directive du Conseil de l'Union concernant le

directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE. La France présidera le prochain G7. Le Président de la République se préoccupe lui-même de l'organisation de ce sommet en se rendant sur place, à Biarritz. Nous souhaitons qu'il s'active aussi fermement sur cette question.

C'est un signal encourageant. Nous le constatons, les positions des États évoluent en fonction de leurs intérêts propres. La réforme de la fiscalité américaine de décembre 2017, destinée à attirer les actifs les actifs incorporels et les bénéfices sur son sol en les rapatriant des paradis fiscaux et à sécuriser l'assiette imposable, en est l'expression. Nous ne pouvons que soutenir votre démarche ; c'est une avancée que nous

Pourtant, mon premier amendement avait pour objet le versement d'une part des résultats de la taxe perçue au titre de l'article 299 nouveau du code général des impôts au Fonds d'aménagement numérique des territoires, le FANT.

résulte de l'activité économique numérique réalisée en France et, par conséquent, de l'accès généralisé aux outils de communication électronique en très haut débit sur notre territoire, objet même de l'existence du FANT la contribution au financement des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux de communications électroniques. Comme indiqué dans le code général des impôts, la réalisation des services taxables est liée à l'accès des utilisateurs aux interfaces numériques, par voie de communications électroniques ; cela implique l'installation de la fibre optique jusqu'au domicile pour tous. L'abondement du FANT, créé pour la bonne réalisation des réseaux de télécommunications envisagés par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, aurait ainsi permis de prolonger le financement du plan France très haut

Sous réserve d'un nouveau dispositif européen en vue d'une harmonisation fiscale substituable à cette taxe, le FANT aurait ainsi pu être abondé postérieurement à 2022, pour la bonne réalisation des schémas directeurs des usages et services en jeu, après la couverture numérique des territoires spécifiée à l'article 33 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Le second amendement que j'avais déposé avait pour objet d'établir les modalités de calcul de la part du produit de la taxe destinée à l'abondement du FANT. Au-delà du prolongement du plan France très haut débit, il est nécessaire d'appréhender le coût particulier d'exploitation dans la durée. Le fibrage de l'ensemble des foyers français, y compris ceux qui sont les plus coûteux à raccorder, bénéficiera à tous, et principalement aux entreprises ciblées par le présent Ainsi, par analogie avec le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, le FACÉ, créé dès 1936 et dont l'objet est le versement de subventions aux collectivités, il serait judicieux et opportun que la taxe versée par les entreprises proposant leurs services numériques

indispensable à la réussite du plan que vous soutenez.

Le texte qui nous est soumis est une bonne réponse, je crois, à la demande de justice fiscale. Il n'est pas acceptable que les entreprises multinationales du secteur numérique soient en moyenne taxées à 9,5 %, alors que les autres, vous l'avez dit, le sont à 23 %.

le voit bien, au travers de toutes les techniques que vous connaissez, dont le fameux sandwich irlandais, ... Le ! ... ou hollandais, tous les bénéfices s'évadent d'abord vers les Pays-Bas, puis vers l'Irlande, et enfin disparaissent aux Bahamas. Le dispositif prévu à l'article 1 s'inspire très largement de celui de la Commission européenne. Il n'est pas parfait, et nous avons à l'esprit qu'il a un caractère l'objectif étant d'aboutir très rapidement à une solution multilatérale ; toutefois, à titre personnel, j'ai des doutes ou des réserves quant au fait que les États-Unis, dans le cadre de l'OCDE, soient

le chiffre d'affaires et non les bénéfices ; je pense que c'est un choix judicieux, car cela évite la neutralisation du dispositif par les conventions fiscales. Certains de nos

Le taux retenu est raisonnable ; il est calqué sur celui qui figure dans la directive européenne. Je ne suis pas favorable aux différents amendements ayant pour objet de le porter à 3,5 %, à 4

Je me réjouis de constater que le Gouvernement, qui, à l'époque, semblait penser la même chose, est aujourd'hui convaincu de la thèse que nous avions défendue et votée en séance budgétaire,

de loi. En l'absence de certitudes sur le plan international, il convient, par prudence, de renvoyer l'extinction de la taxe à un moment ultérieur. Il semble effectivement très ambitieux de considérer que les discussions conduites au niveau de l'OCDE aboutiront d'ici à la fin de l'année 2021. Aussi, mentionner dans l'article une date d'extinction crée une situation ambiguë et contre-productive sur les plans fiscal et législatif. C'est en ce sens que la suppression de cette disposition nous apparaît nécessaire.

d'une taxe nationale, afin de nous donner toute la crédibilité nécessaire à l'OCDE pour obtenir une solution internationale. Vous me permettrez d'être un peu moins confiant que certains dans cet hémicycle sur notre capacité à obtenir un résultat à l'OCDE. Comme qui dirait, chat échaudé craint l'eau froide ... En outre, j'ai pu constater que, en matière fiscale, il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts

au 1 janvier 2020, de manière à leur laisser le temps de développer les outils nécessaires. Je vais citer un exemple. Aujourd'hui, les plateformes effectuent un suivi de l'usage de leurs services, mais, selon les modèles économiques, ce ne vise pas toujours le consommateur et, donc, la valeur créée en France. France. Ainsi, s'agissant des régies publicitaires, c'est l'usage de la plateforme par les annonceurs qui est pris en compte dans le des transactions financières. L'application de la taxe sur les services numériques nécessitera donc, pour les acteurs du numérique, de mettre en place de nouveaux outils, propres à identifier la consultation en France et à y assigner une part de la valeur créée. de la valeur créée. Par exemple, pour une publicité consultée dans toute l'Europe, il faudra, non seulement effectuer le suivi des visionnages en France, mais aussi y assigner une quote-part de ce qui a été payé par l'annonceur. Tout cela imposera donc une refonte lourde des systèmes d'information, qui ne peut pas débuter avant le vote de la loi, puisque la CNIL interdit la collecte de données sans motif légal.

Les recettes, estimées à 400 millions d'euros, soit moins d'un demi-millième du total des prélèvements obligatoires, sont fictives, puisque la France pourrait être contrainte de les rembourser dans quelques années, faute de s'être conformée au droit européen de la concurrence- il y a des précédents. L'assiette retenue, à savoir le chiffre d'affaires, favorisera paradoxalement les gros au détriment des petits et, par conséquent, renforcera la position des géants américains et chinois à l'égard des start-up françaises et européennes, qui ne pourront accroître la dimension de leurs affaires. sans parler des incidences et répercussions fiscales qui viendront grever le pouvoir d'achat des consommateurs français, que l'État s'ingénie, dans le même temps, à stimuler à grand renfort de dépenses publiques ! Pourtant, malgré ces griefs et par excès de zèle « taxateur », nous nous apprêtons à adopter cette

la rétroactivité de la taxe au 1 janvier 2019 n'étant pas la moindre de ses conséquences fâcheuses.

trois mois supplémentaires. Par souci de cohérence, nous modifierions également la date limite pour formuler l'option sur le régime de groupe, prévue dans tous les régimes fiscaux.

Le scrutin est ouvert.